La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 20 mai 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ?

c'est afin d'évoquer, non pas le volet pratique et économique du problème que pose l'émergence de l'illectronisme, mais plutôt son traitement par votre administration, au domaine d'intervention ô combien précieux : l'éducation de nos enfants. Dans le numéro 28

L'équipement informatique et numérique dans les écoles publiques du premier degré est moins généralisé que dans les établissements publics du second degré.

En effet, il est prouvé que la maîtrise de l'informatique fait principalement défaut aux populations les plus fragiles et les plus socialement défavorisées, ce qui n'est pas admissible. Monsieur le ministre, pour que l'école soit une chance pour tous les enfants de la République, l'éducation nationale entend-elle s'attaquer résolument au problème et réduire cette fracture numérique intolérable ? Ne pourrait-elle agir

quelque temps, nous créerons sans doute une agrégation d'informatique, à la suite du Capes. En outre, vous mentionnez l'équipement informatique des écoles, notamment dans les communes rurales. C'est effectivement un grand sujet. En 2017 et 2018, nous avons lancé l'appel à projets « écoles numériques innovantes et ruralité » (ENIR) à destination des écoles rurales, dans le cadre des investissements d'avenir. a permis de financer 3 788 écoles de 3 570 communes. À compter de 2018, c'est un montant total de 20 millions d'euros que l'État a mobilisés dans le cadre des programmes d'investissements d'avenir

de la jeunesse. Monsieur le ministre, la crise que nous traversons met en lumière les fractures éducatives qui durent depuis trop longtemps entre territoires urbains et ruraux. La relance qu'il nous faut préparer peut être aussi l'occasion de révolutionner nos approches et de donner toute sa place à l'éducation en zone rurale, parent pauvre de nos politiques publiques.

quelles suites entendez-vous donner à ces deux rapports pour qu'ils ne restent pas lettre morte ?

quelles mesures comptez-vous adopter pour mieux et davantage prendre en compte le temps de l'enfant, qui, compte tenu des nouvelles pratiques professionnelles des parents, des regroupements scolaires, des temps de trajets ou encore des activités périscolaires, a considérablement évolué ? Ces

elle va entraîner une perte de recettes que le Gouvernement a évaluée à 14 milliards d'euros pour la période 2020-2021. Les communes seront moins affectées que les régions et les départements, elles subiront des baisses de ressources, que ce soit au titre des produits des services, des droits de place, de la taxe de séjour, de droits de mutation ou encore, dans certains cas, des loyers commerciaux.

La mobilisation exceptionnelle des communes face au Covid-19 a également entraîné de lourdes dépenses supplémentaires- je pense notamment aux frais engendrés par la réouverture des écoles. Un certain nombre de communes risquent donc de connaître de réelles difficultés, particulièrement en milieu rural.

de réponse suivants. Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement prête une attention toute particulière à la situation des collectivités territoriales. Vous l'avez dit : les équilibres budgétaires sont parfois remis en cause

par les dépenses déjà effectuées, mais aussi par la baisse prévisionnelle d'un certain nombre de recettes fiscales ; bien entendu, nous les avons toutes et tous en tête. À cette équation budgétaire se sont ajoutés des facteurs de complexification, comme l'impossibilité, durant la période

ces mesures ont bénéficié à plus d'une centaine de communes. Elles restent évidemment à disposition de toutes celles qui le souhaitent. Le Gouvernement s'est aussi attaché à soutenir les collectivités territoriales affectées par un surcroît de dépenses en raison de la crise sanitaire, en contribuant à hauteur de 50 % aux achats de matériel. Comme vous le savez, à la suite de nombreuses observations remontées du terrain, la date de prise en compte des commandes a été avancée, comme l'a annoncé le Premier ministre. Enfin, le Premier ministre a confié une mission au député Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, pour évaluer de manière fine les conséquences financières de l'épidémie sur les structures locales et proposer, en leur faveur, des mesures d'accompagnement. M. Cazeneuve devrait rendre ses propositions dans quelques jours. Il s'attachera bien entendu à les décliner en fonction du niveau de collectivité,

En premier lieu, le 115 nous a fait part d'une hausse assez significative d'appelants et de personnes sans solution depuis le début du mois de mai. À titre d'exemple, le 13 mai dernier, le 115 de mon département, la Seine-Saint-Denis, enregistré 119 personnes laissées à la rue faute de place. En second lieu, en raison de l'arrêt des activités liées au tourisme, les quelque 2 000 places débloquées par les hôteliers en Seine-Saint-Denis ont permis l'hébergement de centaines de personnes vulnérables. Nous nous en félicitons. Mais ces places d'hôtel seront occupées dès la reprise de l'activité. Cette situation soulève des inquiétudes, d'autant que, parmi les personnes hébergées, on compte beaucoup de familles monoparentales. D'autres questions surgissent, comme le manque de visibilité quant au fonctionnement des structures d'hébergement pérennes, qui ont parfois dû réduire fortement leurs capacités d'accueil afin de se conformer aux gestes barrières préconisés. De fait, la place va bientôt cruellement manquer pour assurer à la fois le maintien des personnes mises à l'abri et l'accueil de nouveaux demandeurs, notamment pendant la période hivernale.

le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, ma question porte sur la nouvelle réglementation environnementale 2020, ou RE 2020, qui, au-delà de la révision des exigences énergétiques des bâtiments, doit introduire un nouveau critère lié à la captation et à la séquestration de carbone. À l'issue de la concertation menée, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) recommande une empreinte carbone et un indicateur spécifique pour le carbone dans le bâtiment, mais sans niveau d'exigence pour le stockage.

et biosourcés n'apparaît plus : est-elle écartée ? La seconde concerne l'indicateur de stock de carbone, qui correspond à la masse totale de carbone stockée dans le bâtiment : sera-t-il bien un indicateur réglementaire, assorti d'un seuil ? La parole est à M.

entre le 13 avril et le 1 juin, dans la limite de 84 centimes d'euro pour les masques à usage unique et de 2 euros pour les masques réutilisables. Or, compte tenu de l'urgence, mais aussi des difficultés d'approvisionnement et des délais de livraison, les collectivités territoriales n'ont pas attendu le discours du Président de la République, le 13 avril dernier, pour commander des masques. Par exemple, le conseil départemental de la Nièvre avait anticipé ses commandes pour répondre au plus vite aux besoins de ses agents sur le terrain, mais aussi des

et d'anticipation ! D'autant plus qu'il s'est agi de pallier les imprévoyances et dysfonctionnements de l'État ... À l'heure où le Gouvernement s'appuie fortement sur les élus locaux pour lutter contre le coronavirus et sortir du confinement, le remboursement prévu par l'État n'est pas à la hauteur, ni financièrement ni au regard de la période retenue. Ces conditions de remboursement dégradées pénalisent les collectivités territoriales, dont les finances, déjà tendues avant la crise,

de calcul de la participation de l'État à l'acquisition de masques par les collectivités territoriales, avant de lancer un vaste plan de soutien des finances locales, qui permettra d'accompagner la relance économique à partir des territoires ! La parole

Les dernières années ont été marquées par des retards de paiement de ces aides, largement relayés par la presse ; ils mettent en difficulté de nombreuses fermes engagées dans cette démarche vertueuse. 2019 aura, heureusement, été celle du rattrapage, puisque, aujourd'hui, la plupart des dossiers en retard ont été payés, au prix d'efforts considérables de l'administration et d'une grande patience des agriculteurs. Malheureusement, certaines situations restent problématiques. Ainsi, depuis plusieurs mois, certains producteurs se voient refuser le paiement de leurs aides, voire infliger des demandes de remboursement, sous prétexte qu'ils n'ont pas respecté une règle de rotation des cultures, dont ils n'avaient pourtant pas connaissance. En effet, à cause des retards de paiement, cette règle n'est vérifiée et communiquée que deux à trois ans après la demande d'aide, ce qui ne laisse aux producteurs aucune marge de manoeuvre pour adapter leurs assolements. ces demandes de remboursement sont parfois très lourdes, mettant en péril l'équilibre financier des fermes concernées. Ces producteurs, qui respectent en tout point le cahier des charges de l'agriculture biologique, demandent au ministère la possibilité de s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions. L'annulation de toutes les demandes de remboursement semble un préalable évident, de même que la recherche des moyens administratifs de verser les aides demandées. Un arbitrage ministériel a été rendu sur ce sujet le mois dernier. La profession ne peut s'en satisfaire, puisqu'il n'apporte de solution qu'aux éleveurs et prive encore les céréaliers des aides bio auxquelles ils devraient pouvoir prétendre.

Les producteurs concernés souhaitent tourner la page des retards de paiement, qui ont poussé certains agriculteurs à saisir la justice il y a tout juste un an ! La parole

Du fait des retards de paiement passés, le régime de sanctions n'a commencé à produire ses effets qu'à l'été 2019. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation avait immédiatement prêté attention aux témoignages de nombreux élus de la profession agricole sur le caractère parfois disproportionné des sanctions financières annoncées aux exploitants. Il n'est Il n'est pas souhaitable que des agriculteurs qui s'engagent volontairement dans des pratiques vertueuses pour l'environnement soient sévèrement pénalisés pour des erreurs minimes. D'autant que ces erreurs ont été accentuées par des retards d'instruction

sur les campagnes passées, tout en restant en conformité avec le cadre prescrit par les règlements européens. Ainsi, pour les campagnes de 2015 à 2018, qui ont subi un retard d'instruction, il est notamment prévu que les sanctions soient allégées en cas de répétition d'une même anomalie plusieurs années de suite. Certaines de ces dispositions nécessitent une modification de la réglementation. C'est la raison pour laquelle un nouveau décret, dont la publication est imminente, a été signé par le ministre de l'agriculture : il permettra à l'Agence de services et de paiement, ainsi qu'aux directions départementales des territoires et de la mer, de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures envisagées dès le mois de juin. Les versements ou annulations de pénalités qui en résulteront seront ainsi effectifs dès cet été. Ces nouvelles dispositions apporteront une réponse aux difficultés des agriculteurs visés par des sanctions disproportionnées et garantiront pour l'avenir un régime de sanctions plus juste et plus efficace. Dans l'immédiat et très concrètement, environ 1 500 agriculteurs en bénéficieront dès cet été ; en fonction de la situation de chaque dossier, une part plus importante de leur aide pourra être versée et/ou les pénalités pourront être réduites, parfois, pour plusieurs campagnes simultanées.

notamment dans les Alpes du Sud, où l'évaluation de leur admissibilité est rendue compliquée par le relief et les spécificités locales. En effet, si l'on peut se réjouir des améliorations apportées au dispositif d'évaluation, il est encore nécessaire de faciliter les déclarations des exploitants de perfectionner les modalités du cahier des charges de pâturage pour mieux prendre en compte certains critères. Bien sûr, on peut se féliciter de la reconnaissance, en 2015, des surfaces pastorales peu productives,

La France est-elle en mesure de garantir l'éligibilité de ces surfaces pastorales ? Alors que la pandémie de Covid-19 a stoppé les travaux en cours,

C'est pourquoi la France a farouchement défendu ces surfaces et obtenu leur reconnaissance dans le cadre de la PAC actuelle, principe auquel nous sommes attachés. L'importance de ces zones a aussi conduit le Gouvernement à mobiliser la nouvelle possibilité réglementaire pour étendre la prise en compte de ces surfaces dans trente-huit départements.

le ministre de l'agriculture a lancé, comme vous l'avez indiqué, un travail avec les professionnels pour faciliter et sécuriser la gestion de ces surfaces. Une réunion prévue en mars a dû être reportée, compte tenu des mesures de confinement ; elle sera reprogrammée prochainement, pour que ce travail puisse avancer. La bonne mise en oeuvre de la réglementation est essentielle pour sécuriser juridiquement l'admissibilité de ces surfaces aux aides européennes et promouvoir par ce biais le maintien de l'activité pastorale dans les zones concernées.

le code général des impôts prévoit la possibilité pour le comité d'un syndicat de lever les différentes taxes locales en lieu et place de ces contributions budgétaires. Dans ce cas, le produit fiscal à recouvrer dans chaque commune membre au profit du syndicat est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises. La taxe d'habitation revêt, de toute évidence, une importance non négligeable dans les ressources des EPCI sans fiscalité propre. De fait, le montant perçu au titre de la taxe d'habitation s'est élevé en 2018 à 90 millions d'euros. Or la loi de finances pour 2020 a supprimé la taxe d'habitation sur la résidence principale pour 80 % des ménages et gelé ses taux pour les 20 % de ménages restants. En conséquence, bien que les syndicats de communes conservent la faculté de voter le produit qu'ils souhaitent à compter de 2021, l'imposition sera désormais concentrée sur les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises. termes, vous avez fait le choix très clair de faire peser sur deux catégories de contribuables- les propriétaires et les entreprises -les éventuelles augmentations de fiscalité locale destinées à maintenir à leur niveau actuel les ressources des EPCI sans fiscalité propre. Dans un contexte économique et social normal, cette mesure pourrait s'entendre ; mais dans le contexte de déroute économique que connaît la France en raison de l'épidémie de Covid-19, croyez-moi, monsieur le secrétaire d'État, le consentement à l'impôt risque d'être considérablement amoindri : nos entreprises sont exsangues, et les ménages connaissent des situations financières très tendues

; dans le silence des statuts et en l'absence de disposition expresse, le comité du syndicat est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales. Le syndicat dispose de ressources relevant soit de contributions budgétaires des communes, soit d'une taxe additionnelle sur la fiscalité locale- cette seconde possibilité reportant sur le contribuable local,

taxe foncière sur les propriétés non bâties et cotisation foncière des entreprises -en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées. Le taux additionnel applicable et déterminé en deux étapes. le syndicat arrête un produit fiscal global, réparti entre les quatre taxes proportionnellement aux recettes que chacune procurerait à la commune, si l'on appliquait le taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition- la procédure est prévue à l'article 1636 B du code général des impôts. Cette répartition est obtenue en multipliant le produit fiscal recouvré dans chaque commune par le rapport entre, d'une part, le produit théorique que chacune de ces taxes aurait procuré à la commune si l'on avait appliqué le taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition et, d'autre part, le produit total que les quatre taxes auraient procuré à la commune si l'on avait appliqué le taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition- transmettrai tout cela par écrit ... Ensuite, les taux d'imposition sont obtenus en divisant la part du produit de la taxe additionnelle qui doit être perçue dans chaque commune sur les redevables de chacune des quatre taxes par le total des bases nettes correspondantes imposables au profit du syndicat. La suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale conduit à une nouvelle répartition des produits syndicaux entre les contribuables. Pour permettre cette compensation, les taux d'imposition de la taxe d'habitation, y compris le taux des contributions fiscalisées que nous venons d'évoquer, sont gelés de 2020 à 2022 au niveau de 2019. Ainsi, les effets combinés du gel du taux de la taxe d'habitation à son niveau de 2019 et de la non-fiscalisation des contributions syndicales entraîneront un report de pression fiscale sur les derniers redevables de la taxe d'habitation sur la résidence principale jusqu'en 2022 et sur les redevables de la taxe d'habitation afférente aux résidences secondaires et aux locaux vacants,

Dans nombre de départements littoraux, en particulier en Nouvelle-Aquitaine, cette obligation de fermeture s'étendait voilà peu à tous les hébergements touristiques. Dès l'ordre de fermeture, hôtels et campings se sont exécutés. Il n'en a pas été de même pour certains hébergeurs individuels, qui ont continué à louer par l'intermédiaire des plateformes. Cette situation a été et demeure inacceptable pour les métiers de l'hôtellerie : elle apporte une nouvelle preuve de distorsion de concurrence- soit l'absence d'égalité dans la pratique d'une même activité. À l'aune de l'expérience du confinement et des inégalités constatées par endroits, il apparaît essentiel qu'un protocole sanitaire soit imposé à tous les hébergements touristiques, professionnels comme non professionnels. Les hôteliers ont déjà élaboré le leur, qui énonce des prescriptions concrètes sur l'aménagement des espaces, des services de restauration et des prestations extérieures. Afin de garantir son respect, des contrôles seront, à n'en pas douter, menés strictement. En ira-t-il de même pour les hébergeurs non professionnels utilisant des plateformes ? Comment accepter qu'un hébergeur non professionnel puisse recevoir chaque semaine un nombre substantiel de clients et les faire profiter sans contrainte particulière d'équipements comme une piscine, alors que l'hôtelier, lui, sera soumis à à des règles si contraignantes qu'il risque de renoncer à toute mise en exploitation ? Comment accepter qu'un hôtel soit sanctionné pour un manquement à l'application du protocole sanitaire et que, pour un fait identique,

le sénateur, le comportement de certains propriétaires de meublés de tourisme ou de plateformes, qui n'auraient pas respecté les interdictions édictées par les préfets et les maires durant les vacances d'avril ou qui s'affranchiraient des règles applicables à tous.

Nous avons pris des mesures d'urgence qui ont bénéficié au secteur de l'hôtellerie- chômage partiel et prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, pour aller de l'avant sur le chemin de la reprise, nous allons déployer d'autres mesures pour les acteurs du secteur : exonérations de cotisations sociales patronales pour la période de mars à juin assorties d'un crédit de cotisations de 20 %, maintien du chômage partiel jusqu'en septembre, prolongement jusqu'à la fin de l'année du fonds de solidarité, renforcement des dispositifs de prêts garantis par l'État avec le prêt garanti « État saison augmentation de 250 millions à 1 milliard d'euros de l'enveloppe des prêts tourisme de BPI France. Par ailleurs, nous avons obtenu des banques qu'elles proposent le report des mensualités sur douze mois.

et de montagne. Les mesures d'urgence, bien sûr, ont été les bienvenues ; elles ont d'ailleurs été saluées par la profession, avec l'espérance qu'un certain nombre de contraintes soient

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, micro-entrepreneurs : les travailleurs indépendants sont aussi divers que nombreux puisqu'ils représentent près d'un emploi sur dix en France d'ailleurs. L'Insee les désigne non pas comme des travailleurs indépendants, mais comme des travailleurs non salariés, une définition par la négative qui peine à rendre compte de la diversité du phénomène. ont en partage l'absence de lien de subordination, mais aussi et surtout une prise de risque professionnel et personnel qui, dans le contexte de crise sanitaire actuel, les rend beaucoup plus vulnérables à l'arrêt de leur activité.

Je pense par exemple aux auto-écoles de l'Oise partenaires du Pass'permis citoyen, dispositif que j'ai mis en place lorsque j'étais président du conseil départemental et qui a aidé plus 12 000 jeunes à obtenir leur permis de conduire en contrepartie du temps accordé à une association ou à une collectivité.

Ainsi, certains conseils départementaux, comme celui de l'Oise, pionnier dans ce domaine comme dans d'autres, leur ont proposé une aide d'urgence de 500 euros fondée, non plus sur leur compétence générale, aujourd'hui disparue, mais au titre de la solidarité. Pour clarifier les choses, j'ai déposé, avec mon collègue Arnaud Bazin, une proposition de loi permettant aux conseils départementaux d'exercer une action financière et économique de soutien aux entreprises dans le cas d'une catastrophe sanitaire, comme il leur est possible aujourd'hui de le faire en cas de catastrophe naturelle.

aux entreprises les plus en difficulté qui risqueraient de se trouver dans l'impossibilité de régler leurs dettes exigibles à trente jours, notamment leurs charges fixes telles que les loyers, dues au titre des mois de mars et d'avril 2020. de ces entreprises ne parviennent pas à trouver de financement alternatif, notamment des prêts, pour couvrir ces besoins. Les entreprises éligibles au second volet peuvent bénéficier d'une aide complémentaire d'un montant compris entre 2 000 euros et 5 000 euros en fonction de leur situation. Notre objectif est d'éviter des licenciements massifs dans le contexte que nous connaissons. C'est pourquoi le choix a été fait, pour ce second volet, de concentrer les efforts dans un premier temps sur les entreprises qui emploient au moins un salarié. Toutefois, pour tenir compte de la situation critique des entreprises des secteurs qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1 mars et le 11 mai, le second volet du fonds a été élargi récemment aux entreprises sans salarié- ce qui me paraît répondre à votre question -, si leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 8 000 euros.

Le fonds de solidarité est un dispositif d'urgence qui s'ajoute aux autres dispositifs mis en place par le Gouvernement depuis le début de la crise sanitaire, notamment le report des charges sociales et fiscales, les dispositifs ciblés d'exonération pour certains secteurs récemment annoncés, les prêts garantis par l'État, l'accélération du remboursement des crédits d'impôts et de TVA ou encore la faculté d'octroyer des remises d'impôts. Les entreprises qui répondent aux conditions d'éligibilité au fonds de solidarité peuvent aussi bénéficier d'un report de paiement de loyer, de factures d'eau, de gaz ou d'électricité. Je dois m'arrêter faute de temps, monsieur le sénateur, mais je vous transmettrai des éléments complémentaires relatifs à l'articulation des compétences entre les différents niveaux de collectivités.

et que le chiffre d'affaires a progressé de plus de 4 % cette même année. La direction de Sanofi a en effet décidé d'axer l'essentiel de son activité sur la biotechnique et d'abandonner le secteur de la recherche sur les « petites » molécules. Sanofi se désengage d'axes thérapeutiques majeurs en termes de santé publique- anti-infectieux, neurologie, maladie d'Alzheimer, diabète, maladies cardio-vasculaires. Alors que, en 2008, notre pays comptait onze sites de recherche et développement, il n'en reste plus que quatre aujourd'hui. Dans mon département, le Val-de-Marne, le site de Vitry-Alfortville est touché par la suppression de 124

mettant la France dans une situation de dépendance vis-à-vis des autres pays en termes d'approvisionnement en médicaments, comme nous l'avons malheureusement constaté à l'occasion de cette pandémie de Covid-19. Monsieur le secrétaire d'État, le devenir d'une industrie majeure pour le pays et pour l'indépendance thérapeutique de la France est en jeu. Ces sites de recherche sont en train de disparaître de notre territoire, avec un impact direct sur les sites de production, au profit d'autres pays comme la Chine ou l'Inde. Monsieur le secrétaire d'État, qu'entendez-vous faire

compte tenu de son empreinte industrielle dans notre pays- il compte 34 sites et emploie 25 000 salariés -, Sanofi, septième groupe pharmaceutique mondial, fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement, notamment des services du ministre de l'économie et des finances qui m'a demandé d'apporter des éléments de réponse à votre question. En matière de vaccins contre le Covid-19, le Gouvernement a récemment rappelé l'entreprise à ses obligations, en soulignant que ce vaccin devait être accessible à tous sans discrimination. Depuis, l'entreprise a fort opportunément précisé ses intentions.

notamment pour les batteries ; nous devrons le faire pour le médicament. Le Gouvernement y travaille avec l'ensemble des acteurs du secteur. À n'en pas en douter, le groupe Sanofi trouvera toute sa place dans cette stratégie que l'on pourrait qualifier de souveraineté industrielle. Cela étant dit, en réponse à vos inquiétudes sur l'évolution des effectifs consacrés à la recherche et développement de Sanofi en France, il nous semble important de souligner que la France reste au coeur de la stratégie de recherche et développement du groupe Sanofi puisque 5 000 salariés y travaillent, soit 40 % des effectifs mondiaux. La recherche et développement de Sanofi en France représente ainsi 2,3 milliards d'euros en 2019, soit 35 % de la recherche mondiale du groupe, ce qui correspond, peu ou prou, à la part de masse salariale que je viens La recherche et développement est par nature un domaine qui nécessite une grande réactivité, et il n'est pas anormal qu'une entreprise comme Sanofi réajuste en continu ses priorités au regard de l'évolution de la médecine, mais aussi au regard des compétences dont elle dispose. En Île-de-France, plus spécifiquement dans le Val-de-Marne, le site de recherche et développement et de production de Vitry-sur-Seine a ainsi bénéficié de plus de 300 millions d'euros pour en faire un site de référence dans le domaine très prometteur des biotechnologies de la bioproduction de médicaments, axe prioritaire du comité stratégique de filière des industries et technologies de santé. L'État soutient aussi l'émergence du campus dédié à la bioproduction dont Sanofi est le pilote. Il permettra de doter la région Île-de-France d'un centre de formation digitalisé sur les métiers de la bioproduction.

la justice est le droit du plus faible, alors elle doit devenir une réalité pour nos concitoyens qui sont mis contre leur gré dans des situations d'injustice. Il en est ainsi, dans certains cas, en matière d'héritage. En effet, il arrive que, à la suite du décès de l'un de leurs parents, des enfants réclament leur part au parent survivant. Dans une telle situation, celui-ci peut être conduit à vendre certains de ses biens, comme une voiture ou une maison. maison. Pour faire face à cette situation, différentes possibilités sont prévues par le droit. Les époux peuvent choisir le régime matrimonial de la communauté universelle en intégrant une clause d'attribution intégrale au survivant. Ils peuvent également opter pour la donation au dernier vivant. Dans ce cas, le conjoint survivant récupère par exemple la quotité disponible. Toutefois, il est utile de préciser que la part de cette quotité dépend du nombre d'enfants, et peut donc être très réduite. Par ailleurs, cela entraîne des frais notariaux nécessairement pénalisants. En effet, si la somme à acquitter peut sembler dérisoire pour certaines familles, elle ne l'est pas pour d'autres qui ont parfois du mal à boucler leurs fins de mois. Or, dès lors que le patrimoine a été constitué par les deux parents, il n'est pas juste que les successibles puissent demander leur part avant le décès du parent survivant. C'est pourquoi, afin de protéger ce dernier, il conviendrait de modifier le droit actuel pour faire de la clause au dernier vivant le principe de droit commun. Cette mesure permettrait d'éviter aux parents de devoir se rendre chez le notaire, et les protégerait du comportement des enfants, comportement qui les contraint parfois à se séparer de leurs biens.

Par conséquent, je souhaiterais connaître les pistes envisagées par le Gouvernement pour pallier cette difficulté soulevée par de nombreux Français. La parole

La loi du 3 décembre 2001 a déjà fait du conjoint survivant un héritier légal de premier ordre ; en l'absence de testament, il vient à la succession, aux côtés des enfants du défunt, et reçoit, soit le quart de la succession en pleine propriété, soit l'usufruit de l'intégralité de la succession, le reste revenant aux enfants. Si le défunt souhaite l'avantager de façon plus importante, la loi du 23 juin 2006 lui a permis d'en faire un héritier privilégié. Ainsi, le conjoint défunt peut lui laisser jusqu'au quart en pleine propriété du patrimoine, et trois quarts en usufruit. Le conjoint survivant peut alors jouir de l'ensemble du patrimoine successoral, et s'il ne souhaite pas une propriété partagée avec les enfants, il peut demander que son usufruit soit converti en rente viagère. Cette faveur faite au conjoint survivant peut-être mise en oeuvre très simplement, et à un coût réduit, voire nul- ce qui me paraît répondre à l'une de vos interrogations soit par le biais d'une donation au dernier vivant passée devant notaire, donation dont les frais sont fixes et encadrés par l'État, soit par le biais d'un simple testament, qui est gratuit. J'ajouterai que la loi fiscale est très avantageuse pour le conjoint survivant comme pour le partenaire pacsé, puisqu'ils sont complètement exonérés de droits de succession. Aller plus loin dans la faveur faite au conjoint survivant comme vous le proposez ne nous semble justifié ni d'un point de vue juridique ni au regard des évolutions de la société : renforcer les droits du conjoint, c'est inévitablement porter atteinte aux enfants, notamment à ceux issus d'une précédente union. Lorsque les enfants sont communs, l'atteinte à leur droit pourrait être considérée comme tolérable, puisqu'ils récupéreront le patrimoine successoral au décès du deuxième parent. En revanche, les enfants non communs n'hériteraient pas du conjoint survivant, et ils perdraient alors définitivement tout héritage si le conjoint hérite en premier. Il n'est donc pas envisagé à ce stade d'accroître encore davantage les droits successoraux du conjoint survivant, déjà très favorisé par la législation actuelle. Cela serait source d'un déséquilibre trop important au détriment des enfants, actuellement protégés par la réserve héréditaire. héréditaire. Le rapport sur la réserve héréditaire remis à la garde des sceaux le 13 décembre dernier par un groupe de travail constitué d'universitaires et de praticiens du droit étudie cette question et permet de nourrir la réflexion sur l'évolution du droit en la matière. Mme la garde des sceaux et ses services restent à votre disposition pour échanger sur ces préconisations.

les remplacer par une contribution de vie étudiante et de campus. Cette contribution permet de soutenir des étudiants, qu'ils soient boursiers ou non, notamment en matière de santé ou de vie étudiante.

et j'ai essayé de faciliter au maximum leur accès. Ces derniers mois, la question de la précarité étudiante a pris un tour plus prégnant encore du fait de l'épidémie de Covid-19.

Dès la fin du mois de mars, la contribution de vie étudiante et de campus a été libérée, soit un montant de plus de 139 millions d'euros cette année, pour que les établissements et les Crous puissent répondre aux besoins matériels quotidiens les plus urgents des étudiants, qu'il s'agisse de répondre à des besoins alimentaires, de les aider à acquérir un ordinateur ou à étendre leur forfait de téléphonie pour assurer la continuité pédagogique.

en charge par le chômage partiel. Cette aide ouverte à l'ensemble des étudiants est accessible de manière simple par voie dématérialisée. J'ai également annoncé que nous gèlerions les frais d'inscription pour la rentrée, et nous sommes en train de travailler à la mise en à la mise en place de mesures spécifiques de façon à garantir que l'accès à l'enseignement supérieur ne soit pas un privilège, mais reste ouvert à l'ensemble de notre jeunesse, y compris celle des classes moyennes qui ne bénéficient pas d'aides par ailleurs. La parole est à Mme Marie Mercier,

ma question porte sur le déroulement des examens et concours dans l'enseignement supérieur durant la crise que nous traversons. Ceux-ci font l'objet de vives inquiétudes relatives au respect de l'égalité des chances des étudiants qui s'y présentent, ainsi que de la préservation de la santé et de la sécurité des usagers et des fonctionnaires. En ce qui concerne les classes préparatoires, si l'organisation des épreuves écrites semble bien se dérouler, des incertitudes subsistent concernant l'hébergement des concurrents, notamment en Île-de-France, en raison de la fermeture des internats. Des négociations sont en cours avec les Crous, mais des solutions restent à trouver. Ces questions d'intendance se posent également pour l'organisation des épreuves écrites en outre-mer, où la « mise en loge » des élèves, c'est-à-dire l'isolement en raison du décalage horaire, est remise en question. La situation est plus alarmante pour les concours de première année commune aux études de santé (Paces), dont le ministère a imposé que la deuxième moitié soit maintenue malgré l'épidémie.

comment garantir la sécurité du millier de candidats et organisateurs réunis une journée entière en un lieu clos ? Enfin, d'une manière générale, les établissements sont en attente de directives claires concernant le traitement à réserver aux étudiants dits à risques, ou encore présentant des symptômes du coronavirus

remercie de votre question qui me permet de valoriser le travail exceptionnel qui a été réalisé par les établissements et par les services des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ces dernières semaines.

et le maintien de l'équité du traitement des candidats. Dès le 24 mars, un comité opérationnel de pilotage interministériel consacré à l'organisation des concours et des examens a été constitué, placé sous la direction de Caroline Pascal, doyenne de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Plusieurs annonces ont été faites, et chaque candidat a été informé individuellement des modalités de passage de ses épreuves. La première décision, annoncée le 15 mars, a été la limitation, à titre exceptionnel, et pour cette année seulement, du nombre de concours et des rassemblements qu'ils occasionnent. Il a ainsi été retenu que l'entrée dans l'enseignement supérieur se ferait sur dossier et sur la base du contrôle continu uniquement. Après des consultations avec l'ensemble des établissements, nous avons déterminé les concours et examens qui devaient être maintenus pour des raisons d'équité, notamment les concours d'entrée dans les grandes écoles. Le 17 avril, nous avons annoncé que les épreuves se dérouleraient entre le 20 juin et le 7 août dans le respect scrupuleux des normes de distanciation sociales et des exigences sanitaires. Dans plusieurs cas, il a été également décidé que les concours écrits ne seraient exceptionnellement pas accompagnés d'épreuves orales cette année. Pour ce qui concerne les études en santé, nous avons annoncé le 26 mars que le concours d'entrée en deuxième année serait organisé à partir de la troisième semaine de juin. Nous accompagnons les établissements, notamment celui de Toulouse que vous mentionnez, afin que les choses se passent le mieux possible pour les étudiants. Nous avons préparé un protocole sanitaire qui a été validé la semaine dernière par la mission présidée par Jean Castex et par le ministère des solidarités et de la santé. Les équipes du ministère, les établissements et les rectorats sont mobilisés pour mettre en oeuvre ce protocole qui a été publié. Je comprends évidemment toutes les interrogations suscitées par ces nombreux changements, mais je tiens avant tout à saluer l'engagement des établissements et des centres de formation pour informer et accompagner tous les candidats dans cette période exceptionnelle.

la ministre de la transition écologique et solidaire, puisqu'elle porte sur l'enjeu que représente le sauvetage du capillaire ferroviaire pour le fret agricole et alimentaire. Le fret ferroviaire est un levier majeur de la compétitivité des entreprises de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Il permet l'irrigation des territoires et représente un atout incontestable dans la transition vers une mobilité plus propre et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Responsable de seulement 0,4 % de ces émissions, il permet d'éviter cinquante camions sur les routes par train chargé et représente un outil précieux pour l'atteinte des objectifs ambitieux fixés par la loi relative à l'énergie et au climat du 8 novembre 2019. doit son succès à sa capacité à être au plus près des outils industriels grâce à son réseau capillaire de 4 200 kilomètres. Or, alors que certaines lignes sont déjà fermées pour des raisons de sécurité, près du quart de ce réseau est aujourd'hui menacé. Ce sont désormais des travaux de remise en état qui s'imposent afin d'en assurer la pérennité. À ce jour, le maintien en état des lignes capillaires ne fait l'objet d'aucun plan national concerté et financé. Les opérations, réalisées sur demande de SNCF Réseau, se font au coup par coup, et le plus souvent dans l'urgence, ce qui rend les coûts d'autant plus importants. Les chargeurs sont mis à contribution,

vous prient d'excuser leur absence et m'ont chargée de vous répondre. Le développement du fret ferroviaire constitue effectivement un enjeu majeur pour le monde agricole, et la préservation des lignes capillaires de fret est un facteur indispensable pour y parvenir. Le secteur agricole, tous domaines d'activité confondus, représente près d'un tiers de l'ensemble du tonnage transporté sur ces lignes. Il existe bel et bien un plan national concerté et financé pour le maintien des lignes capillaires de l'État et SNCF Réseau ont engagé une démarche consistant à travailler, ligne par ligne, avec l'ensemble des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et les chargeurs, pour définir les conditions de leur pérennité. Depuis 2015, l'État participe ainsi au financement des investissements en matière de régénération et de remise en état de ces lignes capillaires de fret à hauteur de 10 millions d'euros par an, aux côtés de SNCF Réseau et des autres parties prenantes. La participation de l'État représente en moyenne 30 % du coût total de cette régénération. L'ensemble des investissements réalisés depuis 2015 s'élève à 180 millions d'euros. Ils ont porté sur 35 lignes capillaires de au total 885 kilomètres, dont près de la moitié voit transiter des productions du secteur agricole, des céréales en très grande majorité. L'État poursuivra bien sûr ses efforts en la matière. Mon collègue Jean-Baptiste Djebbari en a fait l'une de ses priorités en définissant deux pistes de travail.

États membres. Aujourd'hui, le Gouvernement travaille en étroite concertation avec les acteurs du secteur pour élaborer cette stratégie de développement du fret ferroviaire, comme le prévoit l'article 178 de la loi d'orientation des mobilités. Cette stratégie a vocation à intégrer l'ensemble des mesures nécessaires au soutien du fret capillaire ferroviaire.

Je note malgré tout deux ou trois points positifs, notamment le fait que vous intégriez la possibilité de faire appel, dans le cadre du, au Fonds européen d'investissement stratégique. C'est effectivement une réponse au travers d'un mécanisme financier innovant.

des travaux de réhabilitation du réseau capillaire ferroviaire français. La

Ainsi, l'agence de l'eau Seine-Normandie, dans le cadre de son nouveau programme, a changé les critères d'éligibilité aux aides à l'assainissement individuel. De ce fait, certaines communes ne sont plus éligibles à ces dispositifs, alors que beaucoup d'habitants en auraient grand besoin.

Cette situation est particulièrement critique en zone rurale où le raccordement aux réseaux collectifs est quasiment achevé et où il ne reste que l'habitat dispersé à traiter. Je souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre des mesures

Les onzièmes programmes d'intervention des agences de l'eau pour la période 2019-2024 ont été adoptés à l'automne 2018. Ils répondent à deux priorités du Gouvernement : d'une part, un recentrage des interventions dans une logique de solidarité territoriale d'autre part, la poursuite et le renforcement des interventions en faveur de la préservation des milieux aquatiques, de la biodiversité et des milieux marins. La question des aides à l'assainissement non collectif a été largement débattue lors de l'élaboration de ces onzièmes programmes. Dans un contexte de restriction des moyens à la fois humains et budgétaires des agences de l'eau et afin de cibler davantage les interventions, qui concourent efficacement à la reconquête de la qualité des masses d'eau et de la biodiversité qui y est associée, l'assainissement non collectif n'a pas été retenu parmi les priorités ministérielles. Certains bassins ont ainsi fait le choix d'arrêter le versement des aides à l'assainissement non collectif. D'autres, dont le bassin Seine-Normandie par exemple, ont limité ces aides aux territoires dans lesquels elles sont nécessaires pour assurer le bon état des masses d'eau ou relèvent d'une priorité d'ordre sanitaire. Ces solutions, qui résultent des échanges qui se sont tenus au sein des comités de bassin, nous apparaissent comme un compromis pragmatique. Pour le bassin Seine-Normandie, les zones éligibles aux aides à l'assainissement non collectif sont dorénavant le littoral,

La prochaine commission des aides de l'agence de l'eau qui se réunira en juin va d'ailleurs examiner le dossier d'attribution d'une aide, qui s'élève à environ 350 000 euros, pour la réhabilitation de 58 installations d'assainissement non collectif dans la commune de Chevannes-Changy. Par ailleurs, les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation ou de réhabilitation de leurs équipements d'assainissement non collectif peuvent bénéficier d'autres aides.

ma question s'adresse à la fois à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'action et des comptes publics. Elle porte sur l'urgence de l'indemnisation des propriétaires, devenus malheureusement tristement célèbres, de l'immeuble du Signal à Soulac-sur-Mer. Pour mémoire, ces propriétaires et quelques locataires avaient dû quitter leurs logements sur injonction préfectorale du fait de l'érosion littorale. Depuis 2014, ils s'acquittent donc du paiement d'un loyer pour un autre logement, de l'assurance, des charges de copropriété et, pour certains, du remboursement

et que le Sénat s'est prononcé à trois reprises à la quasi-unanimité. Un an et demi plus tard, les victimes ne connaissent toujours pas les modalités de mise en oeuvre

C'est en leur nom que je vous demande des explications et un calendrier. La parole

milité pour faire adopter un régime d'indemnisation pour les propriétaires de cet immeuble menacé par le recul du trait de côte. Avec l'ouverture de crédits dans le cadre de la loi de finances pour 2019,

Par conséquent, il existe un risque juridique élevé si l'on autorise l'acquisition de ces biens à des montants plus favorables pour chaque propriétaire, et ce malgré les dispositions de la loi de finances pour 2019, qui ne créent pas un cadre pour l'indemnisation, mais se limitent à l'ouverture de crédits dans la mission « Écologie on ne peut pas exclure l'hypothèse qu'un juge assimilerait cette indemnisation à une libéralité. Monsieur le sénateur, le Gouvernement n'entend évidemment pas revenir sur le vote du Parlement, veut seulement s'assurer que sa volonté sera bien mise en oeuvre, et ce dans les meilleures conditions de sécurité juridique. Les copropriétaires du Signal pourront alors bénéficier d'une juste indemnisation. Au-delà des biens déjà affectés par le recul du trait de côte, le ministère de la transition écologique et solidaire travaille

Deux régions, dont la mienne, les Hauts-de-France, ont ainsi commencé à mener cette expérimentation pour une durée de trois ans, jusqu'à fin 2021. Parallèlement, un rapport remis au Gouvernement en septembre 2019 propose d'accélérer et de simplifier les procédures obligatoires préalables à une implantation industrielle. Le préfet peut ainsi choisir entre une enquête publique et une simple consultation électronique, ce qui marque, une fois de plus, la volonté de s'affranchir des acquis en termes de participation citoyenne, une partie de ce public n'ayant pas la possibilité de répondre à une enquête sur internet. J'en veux pour preuve les travaux de l'actuelle mission d'information du Sénat sur la lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique. En effet, comme l'a rappelé en 2019 le Défenseur des droits, Jacques Toubon- celui-ci a d'ailleurs été auditionné hier par ladite mission -, la dématérialisation à marche forcée des services publics se résume, pour certains citoyens, à un recul de leurs droits, en raison de la disparition de ces services sur certains territoires. Cela vaut, par extension, pour le service de l'enquête publique. Ces phases obligatoires de consultation des citoyens sont de plus en plus considérées, à tort, comme une perte de temps, un frein à la croissance et à la compétitivité. Or elles constituent un dispositif essentiel au service de la démocratie locale, au coeur du fonctionnement de la démocratie participative, et le meilleur moyen de faire remonter aux décideurs le véritable ressenti le véritable ressenti du terrain grâce au commissaire-enquêteur, qui conduit son enquête de manière totalement indépendante. La dématérialisation de l'enquête publique se ferait au détriment du présentiel et ne ferait qu'accroître les frustrations, les incompréhensions et les risques de contentieux. Pourriez-vous assurer les populations du maintien de l'enquête

m'a demandé de vous rassurer et de vous confirmer que l'enquête publique demeure bien le dispositif de référence en ce qui concerne la participation du public pour les projets soumis à évaluation environnementale. Sur les recommandations du rapport du député Guillaume Kasbarian, que vous évoquiez dans votre intervention, le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique prévoit, en effet, la possibilité d'adapter les modalités de la participation du public applicables aux autorisations Seuls les projets ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale sont concernés par ces dispositions. La consultation du public sur ces projets pourra être adaptée par décision de l'autorité administrative

en application de la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite loi Essoc, vise de manière plus large les projets soumis à autorisation environnementale. L'enquête publique est remplacée par la participation du public par voie électronique, comme vous l'évoquiez, à la stricte condition que le projet ait donné lieu à une concertation préalable avec garant.

Toujours est-il que les dispositifs existants sont conformes aux textes qui régissent la participation du public. Ils respectent notamment la convention d'Aarhus, les directives européennes et l'article 7 de la Charte de l'environnement. La procédure par voie électronique offre des garanties au public : ainsi, les citoyens peuvent toujours demander à avoir accès à un dossier sur support papier. sur support papier. C'est aussi au regard de l'importance de la dimension présentielle de la participation du public que les délais de ces procédures ont été gelés dans le cadre des ordonnances relatives à l'urgence sanitaire liée à l'épidémie

Ces frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie sur prescription médicale, et dans un certain nombre de situations : hospitalisations, traitements ou examens pour des patients qui sont atteints d'une affection de longue durée ; traitements ou examens en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle ; lorsque l'état du patient nécessite d'être allongé ou sous surveillance en cas de trajet de longue distance ou de transports en série pour un même traitement. L'ambulance bariatrique est spécialement équipée pour des personnes de très forte corpulence ou en situation de handicap, qui nécessitent un équipage de quatre personnes, voire davantage, et un brancard deux fois plus large. large. Pour ce type de transport, le remboursement s'effectue uniquement sur la base d'un transport habituel, ce qui ne couvre pas l'ensemble des frais de transport. À chaque déplacement, le reste à charge pour le patient est très élevé et peut parfois atteindre plusieurs centaines d'euros, ce qui rend la situation

grâce aux plans obésité qui ont été mis en place ces dernières années. Dès 2013, les 37 centres spécialisés de l'obésité ont été équipés d'une ambulance bariatrique pouvant transporter les patients avec les besoins spécifiques liés à cette pathologie. La volonté d'améliorer la prise en charge de ces patients a été réaffirmée dans la feuille de route obésité pour les années 2019-2022, qui prévoit notamment de renforcer la structure et la lisibilité de cette offre de transport dans chaque région. Cependant, le Gouvernement a bien conscience de l'insuffisance de l'offre actuelle et des difficultés d'accès à ces prestations, en raison notamment des suppléments facturés aux patients lorsqu'ils doivent faire appel à des transporteurs privés ou qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Pour assurer une prise en charge à la fois pérenne et adaptée sur l'ensemble du territoire, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a inscrit l'amélioration de la prise en charge des transports bariatriques, via la prise en compte des équipages ou des équipements supplémentaires nécessaires dans la tarification, parmi les orientations qui cadrent les négociations conventionnelles en cours entre les représentants des transporteurs sanitaires et l'assurance maladie. Au terme de ces négociations,

santé. Monsieur le secrétaire d'État, j'ai déposé cette question, à laquelle j'associe mon collègue Jacques Genest, le 27 février dernier. Depuis, l'épidémie de Covid-19 a fondu sur notre pays et a fait vaciller bien des croyances. Mais elle a aussi prouvé la justesse de certains constats : la crise sanitaire a ainsi confirmé la nécessité de donner à l'hôpital d'Aubenas la fonction dite « support ». Au plus fort de la crise, cet hôpital aurait pu jouer un rôle majeur, notamment en termes de dépistage. habitants, l'Ardèche reste aujourd'hui le seul département de cette taille à ne pas disposer d'hôpital support. Quant au bassin de santé de l'Ardèche méridionale, il regroupe 100 000 habitants

inciterait les praticiens à revenir exercer en Ardèche méridionale et contribuerait ainsi à lutter contre la désertification médicale qui affecte notre territoire. Cette solution n'est pas qu'indispensable, elle est aussi réaliste, monsieur le secrétaire les efforts de tous les acteurs concernés préparent cet établissement à jouer ce rôle dans les meilleures conditions : je pense notamment à la construction d'un service des urgences neuf et à celle d'une future maison des internes. Interrogé sur ce sujet le 11 février dernier par mon collègue député de l'Ardèche, Fabrice Brun, la secrétaire d'État Christelle Dubos

Que de longues procédures pour répondre à un besoin aussi bien identifié, alors que les médecins et les élus, au premier rang desquels Jean-Yves Meyer, le maire d'Aubenas, réclament le retour de l'hôpital support

afin de mettre en oeuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins à la fois sécurisés et de qualité. Elle a ainsi garanti une bonne coopération entre les établissements de santé sur un territoire donné. Cette coopération indispensable

à la délimitation des périmètres des GHT, et sur la nécessité de respecter les bassins de vie et les flux de patients en vue de l'élaboration de ces groupements, afin de permettre la rédaction d'un projet médical partagé structurant pour le territoire, et de corriger les inégalités d'accès aux soins. Outre le fait que la période actuelle nécessite que l'ensemble des forces du système sanitaire se focalisent sur la lutte contre le Covid-19- j'en profite pour saluer, à vos côtés, l'engagement des professionnels -, un bilan du fonctionnement effectif des différents GHT, dont le GHT Sud Drôme-Ardèche, reste indispensable avant d'envisager une concertation qui viserait à modifier d'éventuels périmètres géographiques.

sur les nécessaires conclusions et les enseignements qu'il faudrait tirer de la crise, ainsi que sur les décisions qui en découleront. Je pense qu'il y aurait là une décision sage, qui permettrait de renforcer le maillage sanitaire dans un département de l'Ardèche qui en a grandement besoin. La parole

112 services d'aide à domicile, dépensant environ 82 millions d'euros pour le soutien des personnes, âgées ou dépendantes, à domicile. Particulièrement endetté, il aura du mal à verser une prime à la hauteur de l'implication de ces hommes et de ces femmes, qui se sont mobilisés avec courage.

d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances [ ...] ». Sans vouloir à l'excès jouer les savants, j'ajoute qu'un arrêt du Conseil d'État de 1994 1994 a porté extension de cette disposition à tous les agents de droit public. À l'instant présent, nous rencontrons une difficulté pour les maîtres de l'enseignement privé,

Comme vous l'avez mentionné, malgré le rappel du dispositif légal en vigueur par la direction de la sécurité sociale, certains employeurs relevant du champ de compétences du ministère de l'éducation nationale continuent de refuser, en pratique, de fournir des autorisations d'absence avec maintien du traitement pour des participations à divers conseils- conseils d'administration, commissions ou représentations liées aux fonctions d'administrateur -, notamment dans le cadre d'organismes de sécurité sociale.

de ce même code dispose très explicitement que « les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances [ ...] ». Cette disposition législative a vocation à s'appliquer tant aux salariés de droit privé qu'aux agents de droit public, conformément à une jurisprudence du Conseil d'État, que vous avez rappelée, datant de 1994. Celle-ci précise que ladite disposition « a pour objet et pour effet de créer au profit de tous de tous les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale le droit de bénéficier des autorisations d'absence nécessaires à l'accomplissement de leur mandat, que ces membres soient des salariés de droit privé ou des agents publics ». L'application aux enseignants de l'éducation nationale, indépendamment de leur statut, par ailleurs que, en contrepartie, les organismes de sécurité sociale « remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions

Malgré l'avancée sur un plan législatif des droits pour les enfants en situation de handicap, les familles et associations de parents se heurtent à une réalité complexe, face à l'insuffisante capacité d'accueil des instituts médico-éducatifs

Comment imaginer qu'un enfant, pour qui l'accompagnement spécifique proposé par les IME est reconnu nécessaire, se retrouve sans autre alternative que d'intégrer un établissement scolaire classique qui lui est absolument inadapté, malgré les dispositifs d'aide en place ? Face à cet enjeu de santé publique et dans le contexte de nécessaire réforme de notre système de santé, à la suite des constats tirés de la crise sanitaire que nous connaissons, il s'avère indispensable d'augmenter la capacité d'accueil des IME, sur le court et le long terme, dans les départements souffrant d'un fort déficit de places, comme c'est le cas de l'Ain.

Concernant la situation spécifique du département de l'Ain, sur laquelle vous m'interrogez, l'offre médico-sociale pour les enfants en situation de handicap se compose en effet de 540 places dans les IME, de 407 places

L'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie de financements complémentaires pour faire progresser cette offre en regard des choix et des projets des familles. Il s'agit d'un budget, à l'échelle régionale, Afin d'incarner et de mettre en oeuvre la priorité que nous accordons à ce domaine, le Président de la République a par ailleurs exprimé une ambition forte lors de la Conférence nationale du handicap du 11 février dernier, visant l'inconditionnalité de l'accompagnement et le respect de la diversité des choix de vie.

solution n'a été trouvée en réponse aux difficultés rencontrées au quotidien. L'offre de places sur le territoire, dont pourra bénéficier le département de l'Ain, constitue naturellement un des volets qui le respect de l'ensemble des choix de vie et besoins de scolarisation des enfants en situation de handicap. Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions que je tenais à vous apporter.

Bien avant la crise sanitaire que nous traversons actuellement et le confinement, la scolarisation de ces enfants était un réel problème, en outre récurrent puisqu'il se répète, malheureusement, à chaque rentrée scolaire. En Moselle, les demandes d'accompagnement pour les élèves en situation de handicap affluent, mais les moyens ne suivent pas. Les nombreux échanges que j'ai pu avoir avec les parents aboutissent au même constat : qu'il s'agisse d'obtenir une place dans un établissement spécialisé ou d'obtenir l'aide d'accompagnants, ils se heurtent à des listes d'attente, qui les laissent totalement démunis et isolés. Le déploiement des maisons départementales des personnes handicapées, chargées du traitement des dossiers et de l'affectation des enfants, reste insuffisant pour répondre à l'ensemble des demandes.

République a lui-même reconnu la gravité de cette situation, lors de la cinquième Conférence nationale du handicap, qui s'est déroulée le 11 février dernier. À cette occasion, il s'est engagé à ce qu'aucun enfant ne soit sans solution de scolarisation à la rentrée de septembre 2020. Il avait également annoncé le recrutement de 11 500 accompagnants des élèves en situation de handicap supplémentaires d'ici à 2022. Par conséquent, madame la secrétaire

C'est ce à quoi le Gouvernement s'est engagé. Les difficultés de scolarisation des élèves en situation de handicap que vous évoquez ne s'expliquent pas seulement par la problématique des accompagnants ou du manque de places. L'accompagnement s'organise ainsi grâce à l'engagement permanent des établissements scolaires à s'adapter aux besoins éducatifs- c'est tout l'enjeu de la loi de 2005 : adaptation de l'environnement aux spécificités des personnes handicapées, en particulier des élèves en situation de handicap -, avec l'appui indispensable du secteur médico-social. C'est cette coopération, cette « ouverture » des murs de l'école aux spécialistes du handicap qui peut rendre la réussite possible. La loi pour une école de la confiance, que vous avez citée, fait entrer le service public de l'école inclusive dans le code de l'éducation. Je mentionnerai la création d'un service dédié dans chaque département, doté d'une cellule de réponse aux familles, et l'accélération du déploiement des unités localisées d'inclusion scolaire (ULIS), ainsi que des unités d'enseignement externalisé, maternelles ou élémentaires, notamment pour les enfants autistes. Aujourd'hui, plus de la moitié des 360 000 élèves en situation de handicap scolarisés bénéficient de l'intervention de 100 000 accompagnants. En 2019, 125 millions d'euros supplémentaires ont été consacrés à leur recrutement et 84 % des accompagnants bénéficient désormais d'un contrat de trois ne travaille sous un dispositif de contrat aidé. Leurs actions pour accompagner sans délai les élèves en situation de handicap seront amplifiées à la rentrée de 2020,

les problèmes de scolarisation de ces enfants, il est urgent et impératif que des solutions soient enfin apportées, et ce dès le mois de septembre prochain. La parole

les familles qui en ont les moyens constituent des équipes de spécialistes autour de leurs enfants, afin qu'ils aient une chance de progresser et, parfois, de pouvoir à nouveau intégrer un cycle dit normal. Cet accompagnement de tous les instants est épuisant, physiquement, moralement et financièrement. Lorsqu'elles ne le peuvent pas financièrement, les familles doivent rentrer en France, avec toutes les conséquences que cela implique au niveau de la scolarité des autres enfants et de la situation professionnelle des parents, et sans certitude d'obtenir une place pour l'enfant.

Madame la secrétaire d'État, quelles mesures concrètes peuvent être mises en oeuvre pour aider ces familles et faire en sorte que tout enfant en situation de handicap ou « dys » soit accompagné et pris en charge, qu'il réside en France ou à l'étranger.

Cet investissement en France sera conjugué avec une action pour mieux réguler la qualité et les financements des établissements belges, car, sur ce sujet aussi, nous avons un devoir de qualité. Un travail de conventionnement sera engagé en ce sens pour les structures accompagnant les adultes français, comme c'est déjà le cas

Cela paraît évident, mais, en fait, notre système n'est aujourd'hui pas structuré pour répondre à cette exigence d'accompagnement. Nous poserons des leviers concrets, avec un numéro unique pour toutes les personnes en grande difficulté afin de lutter contre ce risque d'errance et la mise en place, dans les territoires, de communautés d'acteurs en charge, ensemble, de les accompagner. Nous réussirons si État, collectivités et acteurs de l'accompagnement unissent leurs forces. La crise a suscité spontanément ces coopérations, si essentielles.

de leurs besoins de base. Depuis le 5 novembre 2019, la carte ADA, qui permet aux demandeurs d'asile de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), est devenue une simple carte de paiement sans possibilité de retrait d'argent liquide ni d'achat d'achat en ligne. Selon différentes associations, cette nouvelle carte est totalement inadaptée à la situation des demandeurs d'asile. Privés de liquidités, ils verraient se multiplier de nombreux obstacles, et ce plus particulièrement en zone rurale, comme à Ferrette, dans le département du Haut-Rhin. En effet, il n'est pas toujours aisé de trouver des commerces où il est possible de régler par carte bancaire, ou sinon seulement au-delà de montants incompatibles avec les faibles ressources dont disposent les demandeurs d'asile. De nombreux commerces de proximité tels que les boulangeries, La Poste, les transports, mais aussi les cantines scolaires leur sont ainsi rendus inaccessibles. Leur accès au réseau solidaire et d'entraide est également fragilisé, puisque ces acteurs ne sont généralement pas équipés de terminaux de paiement électronique. Le mécanisme du, censé pallier le défaut d'accès à des liquidités, semble, lui, ne pas fonctionner, et, quand il fonctionne, il produirait des effets stigmatisants. La Commission nationale consultative des droits de l'homme considère que le fait de ne pas permettre aux demandeurs d'asile de disposer librement des ressources qui leur sont allouées porte atteinte à leur dignité. Elle rappelle que l'État doit leur assurer un niveau de vie digne qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. En conséquence, quelles mesures envisagez-vous pour permettre aux demandeurs d'asile de disposer d'un minimum de liquidités et préserver ainsi les solidarités fragiles durement construites au sein des territoires ?

pour demandeur d'asile serve à d'autres fins que celles d'assurer des conditions de vie décentes aux demandeurs d'asile. C'était bien l'objet de cette carte de paiement lorsqu'elle a été mise en place. D'ailleurs, avant sa généralisation au territoire métropolitain, cette mesure a fait l'objet d'une expérimentation durant plusieurs mois en Guyane. Aucune difficulté majeure n'a été relevée. Les retours, en particulier ceux des acteurs économiques, ont été positifs et ont montré que la mise en place d'une carte de paiement en lieu et place d'une carte de retrait ne dégradait en rien les conditions de vie des demandeurs d'asile. Dans le cas de Ferrette, la localité que vous évoquez, je tiens à vous informer que le gestionnaire des deux structures d'hébergement pour demandeur d'asile implantées localement s'est engagé à équiper ses résidences de terminaux de paiement, les fameux TPE. En outre, un aménagement important du dispositif a été consenti avec le déplafonnement total du nombre de transactions autorisées. De la sorte, quel que soit le montant de leur transaction, les demandeurs d'asile peuvent continuer à acheter leurs produits de première nécessité dans les supermarchés et les commerces dotés de TPE. de l'intégration (OFII) a d'ailleurs confirmé la possibilité pour les demandeurs d'asile de procéder à de petits achats avec une carte 100 % paiement, 44 % des transactions ayant ainsi porté sur un montant inférieur à 10 euros en novembre 2019. De la même manière, alors que les associations craignaient que les demandeurs d'asile hébergés dans des zones rurales moins bien pourvues en commerces ne puissent disposer librement de leur allocation, il ressort de ce bilan que la carte de paiement a été largement utilisée sur l'ensemble du territoire métropolitain, selon une répartition régionale correspondant à celle des allocataires. La mise en oeuvre de cette mesure continuera de faire l'objet d'un suivi attentif par mes services- je puis vous rassurer, madame la sénatrice en lien évidemment avec les associations accompagnant les demandeurs d'asile. Nous veillerons, le cas échéant, à adapter le dispositif de façon à résoudre les difficultés concrètes qui seraient avérées. La parole

je vous remercie. À l'heure des technologies connectées toujours plus précises, n'est-il pas cocasse que quasiment aucune commune de France ne soit en mesure de connaître le chiffre exact de ses habitants ? Pourquoi ? Parce que se déclarer à la mairie ou notifier son déménagement n'est pas obligatoire en France, contrairement à de nombreux pays. Pourtant, la population française s'avère de plus en plus mobile. Ainsi, plus de 10 % de nos compatriotes changent de lieu de résidence chaque année. c'est une élémentaire pratique de courtoisie et de savoir-vivre, rendre obligatoire le signalement par les habitants de leur arrivée et de leur départ permettrait aux communes de disposer d'une vision juste de leur population afin d'améliorer le fonctionnement et l'évolution de leurs services publics vis-à-vis des aînés, pour les politiques scolaire, périscolaire et d'accueil de la petite enfance, et de n'oublier personne dans les dispositifs qu'elles mettent en place. Par ailleurs, la pratique du recensement ne serait plus nécessaire et les dotations de l'État au budget des communes seraient davantage en lien avec une réalité plus juste et actualisée de la population. Cette déclaration, réclamée par de très nombreux élus locaux, et qui s'avérerait précieuse, monsieur le secrétaire d'État, en matière de lutte contre le terrorisme, pourrait être dématérialisée et commune à l'ensemble des membres d'une même famille. La mairie en accuserait alors réception et pourrait, si besoin, vérifier les déclarations. Un récépissé constituant certificat de domiciliation et valable jusqu'à l'éventuel départ de la commune serait fourni aux nouveaux habitants. Ce document ferait office de justificatif de domicile, nécessaire pour l'accomplissement de toute formalité administrative.

La récente distribution de masques dans de très nombreuses communes de France a démontré, s'il en était encore besoin, que la connaissance précise du nombre d'habitants d'un logement pouvait être utile. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, voici ma question

? La parole est à M. le secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la mise en place d'un nouveau dispositif visant à contraindre l'ensemble de nos concitoyens à se déclarer en mairie, proposition qui a fait l'objet, comme vous le soulignez, d'un débat ici même lors de l'examen du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique. À cette occasion, le Gouvernement avait fait part de ses très fortes réserves, et ce pour plusieurs raisons que je vais rappeler, monsieur le sénateur. En premier lieu, l'exécutif s'est engagé à lutter contre l'inflation législative, notamment à l'égard des collectivités territoriales, et à poursuivre une démarche de simplification et d'allégement des normes et des procédures. Or la mise en place d'une obligation de déclaration de domiciliation en mairie créerait des contraintes et des charges nouvelles pour les communes qui paraissent peu justifiées. En deuxième lieu, la création d'une obligation de déclaration du domicile se traduirait par la constitution d'un traitement de données à caractère personnel et appellerait par conséquent une attention particulière au regard des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés publiques. En effet, le cadre juridique national et européen applicable aux traitements de données à caractère personnel précise que les données sont collectées pour des finalités qui doivent être déterminées, explicites et légitimes. Il en résulte qu'un tel fichier devrait avoir des finalités limitées et conformes à ce cadre juridique et ne pourrait être justifié par son existence même. En troisième lieu, vous présentez cette obligation de déclaration comme un outil permettant d'effectuer un recensement de la population française. Or le recensement effectué par l'Insee est déjà pleinement satisfaisant les données qu'il établit permettent aux communes de disposer d'éléments chiffrés sous forme anonyme afin d'évaluer les caractéristiques de leur population et de gérer en conséquence les services publics locaux, y compris en période de crise sanitaire. Pour l'ensemble de ces motifs, monsieur le sénateur, le Gouvernement reste défavorable à ce dispositif.

de mon département intervenant en faveur des publics précarisés. Depuis 2014, l'Union européenne soutient l'aide alimentaire au moyen de ce Fonds européen d'aide aux plus démunis. En fournissant une aide alimentaire et matérielle à 16 millions de personnes en Europe, ce fonds constitue le principal outil européen de lutte contre la pauvreté. Il finance, en France, un tiers des repas distribués. Or, dans le contexte des négociations du nouveau cadre budgétaire européen pour la période 2021-2027, il apparaît que les moyens dévolus à l'aide alimentaire européenne vont être largement diminués à partir de 2021. Ce fonds, qui était doté d'un budget de 3,8 milliards d'euros pour la période 2014-2020, devrait en effet fusionner avec le fonds social européen FSE+, fonds dans lequel le budget de l'aide alimentaire se chiffrerait entre 2 et 3 milliards d'euros pour sept ans. Si un tel scénario était confirmé, l'aide alimentaire européenne subirait une baisse drastique de ses moyens. Cette aide représente pourtant un socle incontournable pour lutter contre la pauvreté et ses conséquences, en ce qu'elle permet, en plus de mettre à disposition des denrées alimentaires, que se développent autour d'elle d'autres mesures d'accompagnement allant de l'aide à la recherche d'emploi à l'accès à l'éducation, à la culture et aux loisirs. Il s'agit de la réponse irremplaçable, car parfois unique, à l'urgence que vivent des millions de personnes en France et dans toute l'Europe. Le contexte actuel rend d'autant plus impératif le maintien de ces moyens pour permettre aux associations de poursuivre leurs activités de soutien aux populations pauvres et précaires. La crise économique et sociale qui se profile, conséquence de la crise sanitaire mondiale, ne manquera pas d'aggraver la pauvreté et la précarité, de personnes, en France et ailleurs, d'un accès à une alimentation suffisante. Comment le Gouvernement prévoit-il d'agir pour faire de l'aide alimentaire un pilier du FSE+, avec un budget dédié et renforcé, et ainsi lui permettre de continuer à répondre aux besoins immédiats de ces populations ? La parole est

assuré que la protection de nos concitoyens les plus vulnérables est évidemment un volet essentiel de l'action nationale et européenne du Gouvernement pour répondre à l'urgence de la crise. À cet égard, la France a apporté tout son soutien à l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus, le (CRII+),

La Commission européenne a proposé le regroupement de différents instruments financiers à vocation sociale, dont le FEAD, dans un nouveau fonds, le FSE+, lequel serait globalement doté de 120 milliards d'euros sur la période. Lors des prochaines étapes de la négociation, le Président de la République portera avec force la voix de l'Europe sociale, au travers notamment du financement de l'aide alimentaire. Ainsi, soyez assuré que la France est résolue et combative quant au maintien des enveloppes consacrées à l'aide aux plus démunis au sein du budget européen. Au niveau national, et sous l'égide de ma collègue secrétaire d'État, Christelle Dubos, un travail de consultation avec les associations du secteur a été entamé en décembre 2019, sur la base des recommandations formulées par l'inspection générale des affaires sociales. En tout état de cause, les moyens consacrés à l'aide alimentaire seront préservés par rapport à la période actuelle ; c'est un engagement du Gouvernement. Par ailleurs, comme le Président de la République a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, la France persistera dans son choix politique d'utiliser ces enveloppes pour financer des achats de denrées. Soyez assuré de l'attachement sincère de l'exécutif au modèle français de l'aide alimentaire, qu'il ne s'agit aucunement de remettre en cause, mais au contraire de conforter et de pérenniser, d'autant plus dans le contexte d'épidémie que nous connaissons. La parole

Je souligne que les bénévoles de mon département, comme ceux des autres départements français, que ce soient ceux du Secours populaire, du Secours catholique, de la Banque alimentaire, des Restos du coeur, pour pour ne citer qu'eux, attendent le soutien du Gouvernement pour venir en aide à nos concitoyens les plus démunis. J'espère que nous passerons des paroles aux actes et que les moyens seront effectivement au rendez-vous.

de l'Europe et des affaires étrangères. La France métropolitaine a des frontières avec huit pays. De très nombreux Français sont donc concernés les problématiques de la transfrontalité, au premier rang desquels les 360 000 travailleurs frontaliers, notamment en matière d'aménagement du territoire, de mobilité, bien évidemment, mais également de santé et aussi de développement économique, en particulier dans le cas de frontières communes avec des pays particulièrement attractifs, comme le Luxembourg. La région Grand Est en est un parfait exemple, avec la proximité de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg. Des espaces de discussion, d'échanges, d'innovation, de réalisations y ont vu le jour, tels que les fameux Alzette-Belval, unique en son genre, les eurodistricts, ou encore des plateformes numériques comme Frontaliers Grand-Est ou le Centre européen de la consommation. L'État et les élus locaux ont créé et font vivre ces structures afin de mener, à l'échelle des territoires, des projets communs et durables au service de la facilitation de la vie quotidienne des frontaliers. Ces dispositifs sont agiles et mériteraient d'être davantage encouragés par l'État. Les idées et les bonnes volontés ne manquent pas, monsieur le secrétaire d'État, mais des difficultés persistent. Lorsque nous échangeons avec nos voisins sur les questions transfrontalières, nous échangeons principalement avec des gouvernements sur des politiques de codéveloppement dont les sujets relèvent pour beaucoup de l'État. Le sujet de la santé est particulièrement intéressant en la matière. C'est pourquoi nous manquons cruellement d'un interlocuteur national, d'une personne en capacité de négocier d'égal à égal avec les États voisins, de faire travailler ensemble les diverses administrations, de piloter les relations entre le Quai d'Orsay, les divers ministères, les actions de l'État sur les territoires et les collectivités. Les élus et les acteurs locaux qui font vivre depuis des décennies ce dialogue transfrontalier sont en attente d'un engagement fort de l'État, car, malgré une vraie volonté de coconstruction, ces relations peuvent être particulièrement déséquilibrées quand, de notre côté de la frontière, un territoire fragile à la gouvernance morcelée doit négocier avec un État voisin économiquement surpuissant.

La parole est à M. le secrétaire d'État. Madame la sénatrice, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères conduit depuis plusieurs années une stratégie par frontière qui vise, vous l'avez rappelé, à encourager la coopération transfrontalière sous l'égide d'un ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions transfrontalières. Cette coopération transfrontalière est une dimension de plus en plus importante de la construction européenne ; elle est aussi une condition de bon fonctionnement du Marché unique. Ainsi, la stratégie par frontière, en ce qui concerne l'Allemagne, est définie aujourd'hui par le traité d'Aix-la-Chapelle, dont la coopération frontalière est l'un des plus importants chapitres. Nous examinons actuellement la possibilité de conclure un traité similaire avec nos amis italiens, mais nous avons d'autres projets concernant nos autres voisins, avec lesquels nous nous proposons de définir d'un commun accord, et en fonction des spécificités de chaque cas, les orientations et les organes d'une coopération frontalière frontalière renforcée et mutuellement avantageuse, en phase avec les directives et les recommandations de l'Union européenne. Ces orientations diplomatiques doivent naturellement pouvoir s'appuyer sur une bonne coopération des efforts nationaux. C'est ce que nous faisons en étroite relation avec le préfet chargé des questions transfrontalières à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est, par nature, interministérielle. La récente crise sanitaire en effet montré que la dimension frontalière de notre vie socioéconomique devait être pleinement intégrée dans certains des processus de décision nationale, car les interdépendances économiques et sociales qui existent désormais entre la France et ses voisins ne peuvent pas et ne doivent pas, en raison Nous l'avons par exemple constaté avec la question de la libre circulation des personnels français de santé employés chez nos voisins suisses et luxembourgeois. Les conseillers diplomatiques auprès des préfets de région ont ainsi joué un rôle important, afin de coordonner au mieux les décisions mises en oeuvre dans les pays frontaliers, décisions qui n'ont pas été sans incidence pour nos concitoyens concernés. La crise liée au Covid-19 a clairement démontré que nul ne vit et ne peut vivre en vase clos ; nous devons donc réfléchir à la mise en place d'un suivi interministériel encore davantage coordonné et structuré sur ces questions essentielles pour l'avenir de l'Europe. La parole

à M. le ministre de la culture. Ces dernières années, l'enseignement de l'architecture a fait l'objet d'une attention particulière. Tour à tour, plusieurs rapports ont rappelé la nécessité de l'inscrire dans les dispositifs de l'enseignement supérieur et de la recherche et de lui affecter les ressources nécessaires à ses missions

Malheureusement, cette ambition se heurte de plein fouet à la faiblesse- pour ne pas dire à l'inexistence -des moyens budgétaires qui devraient lui être dévolus afin qu'elle puisse réellement prendre corps. Autrement dit, l'écart entre l'ambition théorique affichée et la réalité des budgets qui lui sont consacrés est très important.

De surcroît, les dotations par étudiant selon les ENSA sont très inégales, créant ainsi une rupture d'égalité manifeste entre les étudiants, sans justification aucune. Aucun transfert humain et financier n'a non plus accompagné la réforme précitée, puisque plus de soixante postes administratifs sont restés vacants faute de publication sur la bourse de l'emploi public. Il s'ensuit que les enseignants-chercheurs, accompagnés des agents administratifs volontaires, ont pallié cette défaillance, s'éloignant néanmoins de leurs tâches principales. Cet état de fait ne peut perdurer, vous l'imaginez, sous peine d'épuisement généralisé et de paralysie de l'ensemble des ENSA. À l'instar d'autres établissements de l'enseignement supérieur, la situation patrimoniale s'avère aussi critique pour plusieurs écoles et un investissement massif se révèle donc impérieux pour mieux accueillir les étudiants et les enseignants.

Par conséquent, quels moyens comptez-vous octroyer aux ENSA pour leur permettre d'accomplir pleinement et sereinement leurs missions, lesquelles, dans le contexte crise sanitaire, vont s'avérer encore plus essentielles ? La parole

tend à les rapprocher du modèle universitaire et s'inscrit dans la stratégie nationale pour l'architecture de 2015. Dans la foulée, cinq décrets ont permis de mettre en oeuvre cette réforme : une autonomie scientifique, pédagogique, administrative et financière des ENSA ; un ancrage territorial

La question financière et humaine n'a pas été oubliée, même s'il reste évidemment des chantiers à conduire. S'agissant d'abord de la question des moyens humains, les postes d'enseignant-chercheur ont été sanctuarisés et 65 postes ont été créés en lien avec le ministère Nous avons contribué à la déprécarisation des enseignants-chercheurs avec des transferts de postes de contractuel à titulaire, ce qui a permis un rattrapage à 66 % des titulaires.

Je leur ai annoncé la publication immédiate des postes administratifs vacants en complément de ceux qui ont déjà été publiés en 2019 ou ouverts au concours pour 2020, l'autorisation de recrutement de 149 enseignants-chercheurs en 2020

Cela fait partie des projets sur lesquels nous travaillons. Je voudrais conclure sur une vision prospective, car j'ai également annoncé dans mon courrier du 4 mars l'ouverture d'une réflexion sur l'avenir de la formation et de la recherche en architecture, en lien avec l'évolution de la profession d'architecte.

ministre, vous avez annoncé une série de mesures pour lutter contre ce fléau. Une cellule ministérielle dédiée à ce sujet a été créée et chargée de suivre les affaires qui sont signalées à vos services. Pourtant, dans le cadre du groupe d'études sénatorial Développement économique de la montagne, que j'ai l'honneur de présider, il a été fait état du dysfonctionnement de cette plateforme. En effet, lors d'une audition consacrée aux violences sexuelles dans les sports de montagne, la personne auditionnée, pourtant impliquée dans la défense des victimes, nous a informés des difficultés à trouver le courriel ou le numéro de téléphone permettant de contacter cette cellule. pourriez-vous nous informer des modalités de saisine de cette cellule ? Par ailleurs, pensez-vous que votre ministère a suffisamment communiqué sur son existence pour en faire un outil efficace de lutte contre les violences sexuelles ? Enfin, n'aurait-il pas fallu créer une cellule, indépendante des fédérations et du ministère, pour garantir sa pleine impartialité ? En effet, aucune enquête n'a été mise en oeuvre, comme l'a relevé un article de paru samedi, par la cellule créée concernant des allégations de violences sexistes à l'École nationale de ski et Et si des enquêtes administratives ont été ouvertes, bien que tardivement, l'une est menée par l'ENSA elle-même, dont la gestion du dossier doit nous interroger, et la seconde, confiée à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), porte uniquement sur les conditions d'exercice des éducateurs mis en cause. Elle est donc incomplète, car elle ne vise pas à enquêter sur la gestion des alertes par l'école. De nombreux témoignages existent et ont été portés à la connaissance de votre ministère. Je vous demande d'accorder une attention toute particulière aux victimes, qui vivent un véritable parcours du combattant, quand elles n'abandonnent pas avant le terme des procédures, découragées face à ce qu'elles considèrent comme une impunité. Que comptez-vous faire, madame la ministre ? La

Cette question des violences faites aux enfants, nous nous la sommes beaucoup cachée collectivement. Depuis plus de dix-huit mois et mon arrivée au ministère, cette question des violences dans le sport, je ne l'ai pas évitée. La parole des victimes s'est libérée, et nous avons découvert des faits inacceptables. je ne les accepte pas. Nous avons posé le sujet de manière ouverte et transparente comme jamais, nous l'avons fait en écoutant et en agissant. On m'a critiquée, comme si je me désolidarisais du mouvement sportif, dont je suis issue, comme s'il fallait défendre celui-ci comme un tout, d'un seul tenant. Certes, mon rôle est de défendre le sport, car j'ai été sportive, j'ai été dirigeante bénévole et éducatrice sportive. Je connais les bienfaits du sport pour nos enfants en termes de santé et d'éducation. Le sport mérite d'être encore plus valorisé par notre société. Je veux redire aux éducateurs et aux éducatrices qu'ils sont admirables, qu'on leur fait confiance. Néanmoins, face à ces crimes et à ces délits, j'ai pris mes responsabilités. J'ai réuni tout le mouvement sportif et mobilisé les associations spécialisées. Nous mettons désormais en place des dispositifs nouveaux, comme celui qui vise à contrôler l'honorabilité des bénévoles. Les victimes et les autorités ont dit ce qui ne se disait pas : nous avons créé une cellule de traitement spécifique renforcée qui travaille d'arrache-pied et a été saisie en quelques mois de plus de 150 affaires. Nous avons sécurisé un circuit de traitement et d'information robuste dans les affaires qui font l'objet de plusieurs types de procédures administratives, judiciaires, voire disciplinaires sportives. Cela vaut pour tous nos établissements, nos services centraux comme déconcentrés, nos fédérations et nos clubs. Tous les faits font l'objet d'un contrôle administratif. Tous les faits font l'objet d'un signalement au procureur de la République aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale et tous peuvent amener à des procédures disciplinaires. Aucun cas signalé n'est à l'abandon, cela vaut aussi pour les faits que vous mentionnez à l'École Le ministère s'est saisi des signalements dès le mois de février. Nous aurons connaissance prochainement des résultats des enquêtes en cours. Notre ministère n'est plus aveugle, toute la chaîne des responsabilités est examinée, car cette chaîne, depuis des dizaines d'années, a fauté à tous les étages. C'est pourquoi j'ai aussi missionné une inspectrice générale du ministère pour étudier la manière d'être encore plus efficace en réponse à la détresse des victimes. Elle nous fournira ses premières pistes de réponse en juin. Elles porteront sur le contrôle de l'honorabilité, la formation des éducateurs et la prévention au sein des établissements et des fédérations. Vous me demandez, monsieur le sénateur, si nous pourrions faire mieux.

Mme la ministre des armées. Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur l'accès aux archives historiques. Je souhaite attirer votre attention sur les conséquences néfastes du décret du 2 décembre 2019,

sont de nouveau soumis à une procédure de déclassement longue et fastidieuse. Ces restrictions risquent d'entraîner des délais de communication très longs, voire de rendre impossible l'accès à des archives pourtant communicables de plein droit selon le code du patrimoine. Les chercheurs usagers des archives publiques françaises, en particulier du service historique de la défense, sont depuis peu dans l'impossibilité de consulter des documents postérieurs à 1940 qui devraient être accessibles selon la loi, au prétexte qu'ils ont été tamponnés « secret » lors de leur production.

pour la recherche de la vérité, fondement de la recherche historique, et pour la réputation internationale de la France en ce domaine. En outre, ces restrictions risquent de criminaliser toute personne qui divulguerait des informations contenues dans des archives estampillées « secret défense » qui, depuis des années, voire des décennies, ont été massivement communiquées. Pour toutes ces raisons, de nombreux acteurs, dont un collectif de douze historiens de divers pays,

Je souhaite vous indiquer que le ministère applique la loi et les règles. Les premières règles sont celles de communicabilité posées par le code du patrimoine-

par l'instruction interministérielle n° 1300 de 2011, qui vient appuyer cette protection du code pénal. Ces règles indiquent que communiquer aujourd'hui un document classifié sans démarquage préalable menace la sécurité juridique des lecteurs comme celle des personnels des dépôts d'archives. Cette obligation de protection s'impose à tous et a été rappelée à la mi-juillet 2019 par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Pour appliquer ces règles, il convient de procéder à une déclassification de chaque document revêtu d'une mention de classification, ce qui entraîne, comme vous l'avez souligné, une mise en oeuvre complexe et des délais globalement longs. En aucun cas, le service historique ne ferme des fonds dont la consultation est indispensable au travail de mémoire. Conscientes de la gêne occasionnée dans l'exercice des missions des chercheurs et historiens par la mise en oeuvre de ces instructions, Florence Parly et moi-même avons pris des mesures d'application immédiate. Premièrement, le chef du service historique des archives a été autorisé à prendre des décisions de déclassification sur les documents du ministère de plus de cinquante Seuls les documents classifiés par des autorités extérieures au ministère continuent ainsi à nécessiter un accord exprès du service émetteur.

Désormais, la décision de déclassification sera réalisée au carton. Nous étudions actuellement l'extension de cette procédure de déclassification au carton

Le service interministériel a mis à disposition des archives, mais il s'agit d'archives triées. Pour le reste, si les mesures que vous venez d'évoquer n'étaient pas prises, le travail des historiens pour aller pour aller au bout de la vérité serait entravé. Les premières mesures que vous annoncez sont nécessaires. J'espère qu'elles permettront véritablement aux historiens de travailler dans les meilleures conditions. Nous